Monsieur le président,

politique du scrutin. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, présentée par MM. Rémy Pointereau, Martial Bourquin et plusieurs de leurs collègues.

révolutionnaire en France, car il simplifie considérablement les rapports entre le propriétaire d'un local commercial et son exploitant. Surtout, il constitue un formidable outil pour les nouveaux commerçants,

Pour les entreprises de moins de cinq salariés, il peut même être maintenu de manière dégressive pendant neuf ans. Pour rappel, sont considérées

au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les zones de revitalisation rurale. Cette mesure ne s'appliquerait que dans les intercommunalités à faible densité, à savoir celles qui comptent moins de 20 habitants au kilomètre carré. kilomètre carré. Ce dispositif, qui, d'ailleurs, a déjà été présenté au titre du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, ne peut être accepté parce qu'il n'a pas de rapport avec cette proposition de loi.

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture sont à même de fournir une véritable expertise, qu'il s'agisse de l'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de la consommation des terres agricoles. proposition de loi indique que ces instances seront présentes au sein de la CDAC, avec avis consultatif. Toutefois, les délais de saisine et d'instruction des dossiers ne permettent pas toujours une expertise approfondie. cet amendement, nous proposons donc que le préfet, président de la CDAC, puisse solliciter les chambres consulaires sur un projet d'implantation commerciale en amont de l'examen du dossier par la CDAC. Dans ce cas, la demande du préfet devra être formulée un mois avant l'examen du projet par la CDAC.

À nos yeux, il est préférable d'améliorer la composition du dossier de CDAC par voie réglementaire. Il sera également utile de favoriser à la fois le partage de bonnes pratiques et d'éléments d'interprétation du droit.

volonté : elle affirme la volonté du Sénat et des sénateurs de mener une action déterminée pour la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Il s'agit là d'une question de souveraineté pour nos élus

c'est un vrai plaidoyer pour que les personnes concernées, qui vivent la ville au quotidien, qui vivent le commerce au quotidien, soient au coeur des décisions. Il faut donc absolument le soutenir, et moi, j'y crois ! Mes chers collègues, encore une fois, je veux vous parler de mon pays je veux vous parler d'un petit territoire, comme le vôtre, monsieur le président, où chaque battement de cil de la moindre fourmi prend des proportions extraordinaires. La décision d'ouvrir

cet article, nous souhaitons rendre plus performante l'évaluation des projets d'implantation commerciale, en prenant en compte leurs effets sur les territoires. Aujourd'hui, pour l'implantation

l'on peut douter que ces foncière aient besoin d'économiser 200 000 euros, le principal écueil réside dans les prémices du raisonnement, à savoir le fait que des grandes surfaces seraient de vraies locomotives en centre-ville. C'est parfois vrai et parfois faux : notre groupe de travail a examiné la question avec des urbanistes. Or la progression du commerce d'enseigne dans les centres-villes s'est accompagnée, dans le même temps, d'une contraction du tissu commercial et d'une progression et d'une progression de la vacance commerciale dans ces mêmes centres-villes. Dans ces conditions, nous proposons que l'implantation des grandes surfaces en centres-villes puisse apporter un début de solution à la situation et nous pensons qu'il ne faut pas supprimer

commission des affaires économiques de revenir sur sa position en expliquant pourquoi cet article instituant des moratoires est nécessaire. Il s'agit de donner une base juridique solide à des moratoires locaux déjà existants.

Ces derniers appliquent à nos territoires des analyses statistiques qui ont une valeur relative, car elles ne reposent que sur quelques observations de niveaux d'eau atteints. En conséquence, de nombreux centres-bourgs se retrouvent injustement classés en zone rouge, Ri1, à risque fort, c'est-à-dire inconstructibles non aménageables, et une trop grande étendue des zones d'expansion des crues, Ri3, limite l'étalement de ces bourgs. Si ces plans ont été présentés lors de réunions publiques, les habitants et les élus ne partagent pour autant ni les notes de présentation, ni les documents graphiques, et encore moins les conclusions, souvent inadaptées à la réalité de nos territoires. À long terme, certains de ces classements préparent de manière injustifiée la désertification de nos zones rurales, de nos centres-bourgs, et paralysent la politique de développement de ces communes. Nous ne pouvons plus continuer de nous limiter à une présentation par les services de l'État des des conclusions de cabinets éloignés des réalités locales qui refusent d'intégrer les aspects humains et ne se fondent que sur les résultats de modélisations contestables. Mme Jourda illustre son propos avec l'exemple de certaines communes de la haute vallée de l'Aude situées sur des bassins versants de faible superficie et qui n'ont jamais connu d'aléa de crue centennale de grande amplitude relaté officiellement depuis 2 000 ans. La probabilité concrète d'un aléa majeur avec risque fort est donc inférieure à 1 sur 2 000. Pourquoi ne pas tenir compte des nouveaux aménagements réalisés depuis 1900 qui contribuent à diminuer les risques d'inondations ? Pourquoi imposer des mesures de blocage de l'urbanisation de nos communes qui sont incompréhensibles pour nos concitoyens et nos élus et font oublier la mission première des PPRI, à savoir définir puis accompagner les aménagements que l'État juge nécessaire pour écarter de nouveaux risques ? C'est pourquoi, mes chers collègues, cet amendement vie à rendre obligatoire, lors de l'élaboration des PPRI, la réalisation d'une étude d'impact sur les conséquences conséquences de l'application de ces plans sur l'attractivité économique des communes et sur le risque de désertification des centres-bourgs, étude d'impact à laquelle seraient obligatoirement associés les élus concernés. Quel

explication de vote. Ces cartographies, fournies par l'État et par des cabinets plus ou moins spécialisés, en tout cas plus ou moins imprégnés de la réalité du terrain, sont des données altimétriques.

permettre aux collectivités de bénéficier d'une ressource complémentaire pour mettre en oeuvre la politique que cette proposition de loi supporte ; freiner la consommation de terres qui est un des vrais sujets aujourd'hui ; participer au rééquilibrage des charges entre le centre et la périphérie.

contournant la loi, comme cela s'est déjà vu par le passé, établirait un parking plus ou moins proche de son commerce et plus ou moins

cette surface correspondant déjà à un hypermarché. En outre, l'exonération proposée par la commission conduirait à soustraire à la contribution, pour le seul commerce alimentaire, plus de 11,5 millions de mètres carrés

4,7 millions de mètres carrés, pour un manque à gagner de 56 millions d'euros par an. S'agissant des stationnements, la proposition de la commission, qui conduit à exonérer des parkings d'environ 40 places, n'est pas modifiée. Enfin, le IV de cet

sert essentiellement à abonder le budget de la Société du Grand Paris pour la construction du métro automatique. La taxe sur l'artificialisation ne s'ajouterait donc pas à la taxe sur les bureaux ni à la surtaxe sur les surfaces de stationnement instaurée par la loi de finances pour 2015.

nous craignons des difficultés liées aux principes constitutionnels et communautaires. Il existe en effet un risque de rupture d'égalité entre l'activité de stockage destinée au commerce traditionnel et celle destinée au e-commerce,

tend à donner une valeur législative à l'engagement du Gouvernement en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. Cette méthode est en effet responsable de la perte de 236 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers par jour, ce qui correspond à la consommation d'un département français tous les sept ans. Certaines formes d'artificialisation, tel l'étalement urbain, peuvent participer à la dégradation de la qualité de vie des citoyens de leurs conditions sanitaires. Elles peuvent aussi engendrer un coût important pour les collectivités territoriales, puisqu'une faible densité est souvent défavorable au principe de mutualisation sur lequel repose la gestion des services urbains qu'elles également une perte d'espaces effectivement ou potentiellement disponibles pour la biodiversité, ainsi qu'une perte de ressources agricoles et naturelles. Elle entraîne souvent une exposition accrue aux risques naturels- inondations, glissements de terrain ... Elle est donc synonyme de destruction, de fragmentation et de cloisonnement des milieux naturels. Cet amendement vise à préciser, dans les règles générales d'utilisation du sol, que les actions des collectivités territoriales doivent contribuer à atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette en 2025. Quel est l'avis de la commission La commission considère que cette préoccupation est très largement satisfaite par les éléments législatifs en vigueur, puisque l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme assigne objectifs à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme. Le du 1° de cet article impose, en particulier, « une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels L'amendement proposé est donc en partie satisfait par le droit en vigueur. De plus, il comporte un objectif « zéro artificialisation nette » très volontariste, mais sans doute un peu trop rigide pour s'adapter aux besoins

l'ensemble de notre territoire et non pas seulement les centres-villes et centres-bourgs. L'artificialisation des sols est principalement engendrée par la construction de logements,

Il convient donc d'avoir une approche équilibrée de ce sujet, afin de concilier au mieux la protection des sols et le développement économique. Le code de l'urbanisme encadre d'ores et déjà l'étalement urbain et l'artificialisation des espaces agricoles, naturels et forestiers, par l'intermédiaire des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et des plans locaux d'urbanisme. Plusieurs exigences l'attestent : le bilan de consommation d'espace à dix ans, la fixation d'objectifs de limitation de la consommation future ou l'encadrement des modalités d'ouverture de zones à l'urbanisation en l'absence de SCOT. Des travaux sont toutefois engagés pour aller plus loin, au sein du Comité pour l'économie verte du ministère de la transition écologique et solidaire ou de la mission d'information pour le foncier agricole de l'Assemblée nationale. Il nous semble donc prématuré de fixer un objectif de lutte contre l'artificialisation des sols sans l'intégrer dans ces réflexions globales

M. Alain Fouché. Cet amendement tend à lutter contre la déforestation importée dans les achats de l'État, dans la perspective des engagements de lutte contre l'artificialisation des sols en France et à l'étranger.

La plupart des entreprises privées visées par la stratégie ont déjà des engagements « zéro déforestation » pour 2020. Il existe même des certifications et des démarches certifiées par une tierce partie indépendante permettant de garantir l'absence de déforestation, l'huile de palme- on en parle beaucoup actuellement -, du cacao ou des noix. Nous proposons donc d'instaurer cet objectif pour le secteur public pour 2022, puisque la majorité des achats publics sont effectués auprès de ces entreprises.

Le Gouvernement travaille actuellement à l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée pour 2018. Celle-ci concerne surtout l'impact de certaines productions sur la déforestation à l'échelle mondiale. je vous renvoie au projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, que notre assemblée examinera bientôt et dans lequel les députés ont inséré des dispositions

au même problème. Ne pénalisons pas les entreprises françaises au prétexte qu'on veut résoudre un problème de centre-ville dans des villes moyennes. Il est dommage qu'une si belle proposition de loi soit entachée d'un tel défaut.

gêné par cet article 27, relatif à la question du commerce électronique. Dans sa première version, cet article visait à créer une taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. Outil inapplicable, il aurait posé une légion de problèmes : problème de recouvrement pour les sites étrangers, problème de surcoût à la livraison, problème de mise en cause de La Poste, champion français de la livraison liée au commerce électronique. outre, des échanges en commission ont montré que, sur la base de 0,5 euro par kilomètre, cette taxe aurait engendré des frais de près de 400 euros pour un déplacement entre Lille et Toulouse. Une telle taxe aurait donc littéralement tué le commerce électronique et accru l'enclavement des territoires ruraux, qui ont retrouvé l'accès à des biens et des services grâce au commerce en ligne.

double imposition pour les commerces physiques, coût d'arrêt sur les investissements dans le secteur des entrepôts, lourdes pertes d'emploi et importantes délocalisations. Pour toutes ces raisons,

des centres-villes et des centres-bourgs ? Voulons-nous établir une véritable équité fiscale entre le commerce physique et les géants du e-commerce ? Cet amendement permet de répondre positivement La taxe sur les livraisons du e-commerce permet de lutter contre les externalités négatives provoquées par la multiplication anarchique de ces livraisons : consommation d'énergie fossile, pollution, suremballage ... Elle vise à encourager les géants du e-commerce à implanter davantage

par géolocalisation. Toutefois, pour tenir compte des inquiétudes exprimées en la matière, il est proposé une nouvelle méthode de calcul fondée sur un pourcentage du prix du bien commandé. Le taux de la taxe est ainsi fixé à 1

Je le répète, le dernier entrepôt de stockage ne sera en général situé qu'à quelques kilomètres du consommateur. Pour tenir compte des situations particulières, nous proposons de nouvelles exonérations lorsque le point de livraison est un bureau du service public de La Poste

Quel est l'avis de la commission

modalités ne conduisent donc plus à un montant très variable et parfois très élevé. Subsistent néanmoins trois difficultés. La première tient au calcul de la taxe. Sur ce point, je ne partage pas l'optimisme de l'auteur de cet amendement. En effet, comment garantir la capacité de notre administration fiscale à récupérer les informations concernant la distance parcourue pour la livraison du bien ? En théorie, ces données devraient pouvoir être disponibles ; en pratique, on

qui sont propriétaires des données. Il ne faudrait pas que la taxe soit mise en oeuvre au détriment de nos entreprises, qui cherchent depuis quelques années à surmonter leurs difficultés en développant des activités de commerce en ligne.

agit de façon extrêmement ferme sur le plan communautaire, ainsi qu'au sein de l'OCDE, pour faire adopter des principes qui nous permettent, collectivement, et plus efficacement au plan international, de taxer les opérateurs du numérique de façon coordonnée.

Ce n'est pas une manière de m'en laver les mains ! Je comprends que nos collègues cherchent à trouver des moyens pour financer ces plans. Cela étant, la commission des finances a beaucoup travaillé sur la fiscalité du commerce électronique.

pays. Le nouveau ministre allemand du budget a dit que cela conduirait inévitablement à une fiscalisation des Mercedes et des BMW vendues aux États-Unis.

seulement une orientation, mais aussi les moyens de cette orientation. Si nous ne disposons pas de ressources suffisantes, nous ne pourrons pas alimenter une nouvelle régie des centres-villes, le FISAC.

Et nous rechignerions à taxer ceux qui aujourd'hui deviennent de plus en plus riches grâce au commerce électronique, créant, par effet domino,

? Encore une fois, un peu de volonté, un peu de bon sens ! Et on verra que lorsqu'on veut, on peut ! Eh oui ! Il n'est de vent favorable qu'à celui qui sait où il va

d'être amélioré, affiné, parce que je ne voudrais pas qu'il mette en difficulté des entreprises françaises. Je me pose également la question des entreprises, de plus en plus nombreuses, qui font

le diable se loge dans les détails.

Voilà donc un autre argument, au chapitre de la faiblesse technique. Nous sommes tous d'accord : il faut faire quelque chose pour les centres-villes et les centres-bourgs. Mais il faut se laisser le temps, peut-être, de trouver des outils plus efficaces,

donc de réorienter une partie de l'épargne vers lesdits centres-villes, qui ont besoin d'investissements pour procéder à la rénovation des bâtiments.

à l'obligation de consacrer 20 % de leurs moyens à des investissements dans des opérations situées dans les centres-villes ou dans un certain nombre de zones qui nécessitent ce type d'interventions. Cette disposition figurait dans la proposition de loi initiale. La commission des finances avait décidé d'y renoncer. Nous proposons de la rétablir telle qu'elle était initialement prévue.

D'une part, il méconnaît la réalité de ces sociétés, qui sont souvent spécialisées dans un type d'immobilier spécifique : certaines font plutôt de l'hôtellerie, d'autres des entrepôts, d'autres encore des bureaux, d'autres enfin du commerce, de telle sorte qu'il pourrait être difficile pour une société, vu

dispositif proposé risquerait d'être contre-productif et d'entraîner un effet d'éviction des investissements, d'abord au sein des catégories de « pierre-papier », ensuite et surtout à destination d'autres pays- les capitaux, en effet, sont très mobiles ; or il existe, dans les autres pays européens, le même type de sociétés, mais pas le même type de contraintes.

certaines dispositions, sur le commerce en ligne, ne nous satisfont pas forcément, mais que de réelles propositions, concrètes, sont faites pour les centres-villes et les centres-bourgs.

Tous les matins, quand je me lève, j'interpelle les consciences. Tous les matins, quand je me lève, s'agissant de ce sujet qui nous intéresse, les centres-villes et les centres-bourgs, je plaide pour des actes d'achat conscients.

Mon dernier libraire a fermé, la semaine dernière, en mettant quatorze personnes au chômage, m'expliquant, la larme à l'oeil, que 80 % de ses pertes étaient causées par le commerce en ligne. Pour cette j'ai le droit de dire, j'ai le droit d'éveiller, j'ai le droit de réclamer ! Nous sommes ici pour faire de la politique, pas pour entrer dans des détails. Quand même ! Le détail devient secondaire ; l'essentiel c'est de dire que nous sommes vent debout contre certaines démarches

Le scrutin est ouvert.